sous les réserves d'usage. Comme M. le président du Sénat et MM. les questeurs en ont informé l'ensemble des sénateurs hier, je vous indique que le port du masque est désormais obligatoire dans l'ensemble des salles de réunion et des circulations du Sénat à compter d'aujourd'hui. Il vous est donc demandé, à partir de ce jour, de bien vouloir porter un masque dans l'hémicycle. L'ordre du

l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytosanitaires prescrit le respect d'une distance de sécurité de dix mètres à partir des limites de propriété des riverains pour l'usage de la majorité des produits aujourd'hui utilisés pour lutter contre les les maladies cryptogamiques de la vigne et de l'arboriculture. Le respect de la nouvelle réglementation va entraîner une réelle impasse technique pour lutter contre le fameux mildiou- l'une des principales maladies cryptogamiques de la vigne, très présente en

en Bourgogne, par exemple. Cela représente des difficultés supplémentaires pour les professionnels de la viticulture, déjà fortement mis à mal par les taxes Trump, les effets du confinement et la chute de la consommation. À terme, cette décision pourrait conduire à l'arrachage de plusieurs centaines d'hectares de vignes qui se transformeraient en friches, avant d'être vraisemblablement urbanisés, les

Afin de sortir de cette impasse, certains viticulteurs proposent d'autoriser l'utilisation du cuivre, produit homologué en agriculture biologique, jusqu'à la limite de propriété des riverains pour une période transitoire de quatre ans au minimum, soit jusqu'au 31 décembre 2023.

produits phytopharmaceutiques intègre la prise en compte de distances de sécurité à l'égard des riverains, conformément à la réglementation européenne et à la loi française.

Je rappelle que ces distances peuvent être modulées et complétées dans le cadre des chartes départementales. Comme vous l'avez souligné, madame la sénatrice, les produits de biocontrôle, les produits à faible risque et les substances de base sont exemptés de ces distances.

Certains établissements de l'enseignement agricole, dans le cadre des enseignements optionnels ou facultatifs, proposent un enseignement dit « de pratique professionnelle

qui doit venir en complément des référentiels de formation et répondre aux attentes des élèves accueillis dans les établissements. Cet enseignement

Les objectifs sont le suivi des populations, la participation à la gestion durable des milieux, la création de partenariats avec les acteurs des territoires. Il ne s'agit en aucun cas d'un certificat visant à développer telle ou telle pratique cynégétique, quelle qu'elle soit. La direction générale de l'enseignement et de la recherche va modifier la note de service du 18 juin 2019 relative aux enseignements facultatifs dans les établissements d'enseignement agricole, incluant des préconisations spécifiques pour les pratiques professionnelles en lien avec le bien-être animal. Par ailleurs, une note sera adressée par la sous-direction des politiques de formation et d'éducation aux directions de mon ministère afin que des consignes de vigilance soient données aux responsables en région de la validation des ouvertures des enseignements optionnels en lien avec la thématique cynégétique.

La désertification médicale est endémique en Seine-Maritime. Les responsables des collectivités locales s'arrachent les cheveux pour conserver ou installer des médecins, tandis que nos concitoyens renoncent à certains soins,

pour l'université de Rouen, et seulement trois en 2021. Je crains que cela ne permette pas d'enrayer la désertification médicale ... Le Gouvernement a aussi prévu le recrutement de 400 médecins salariés. Combien sont destinés à la Seine-Maritime et qui décidera de leur installation ? ? De plus en plus de collectivités locales doivent faire appel à des médecins possédant des diplômes étrangers pour améliorer la situation, mais des maires m'ont alertée sur leurs difficultés à faire reconnaître la certification de ces médecins, et le décret qui vient d'être publié, après des mois d'attente, ne rassure pas

La Normandie fait en effet partie des régions de France métropolitaine où la densité médicale est particulièrement faible, avec de grands contrastes selon les territoires. Face à cette situation, plusieurs réponses sont apportées pour renforcer l'accès aux soins

le nombre d'internes en médecine qui entrent en formation à l'université de Rouen s'est accru de 13 % entre 2013 et 2019. Par (CHU) de Caen et de Rouen et les universités de la région soutiennent fortement les dispositifs de post-internat pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes médecins Chaque année, soixante-dix postes d'assistant sont financés par l'ARS, à hauteur de 6 millions d'euros, pour permettre un exercice à temps partagé entre le centre hospitalier universitaire et les hôpitaux périphériques dans les territoires. En Seine-Maritime, près de 300 jeunes médecins sont passés par ce dispositif depuis dix ans. En moyenne, 75 % d'entre eux font ensuite le choix d'exercer dans la région. Les doyens des facultés de médecine mettent également en oeuvre une démarche, baptisée « territoires universitaires de santé », à identifier et à reconnaître, dans les centres hospitaliers, des praticiens hospitaliers qui se verront confier des missions universitaires. Il

C'est dans ce même esprit que le Gouvernement a mis en place le dispositif des « 400 médecins généralistes », qui partageront leur temps entre un hôpital et des consultations dans une zone sous-dense ou exerceront à titre salarié dans un centre de santé. En Seine-Maritime, dix projets sont engagés.

des médecins, hors quartiers prioritaires de la politique de la ville, soit une augmentation de dix-neuf points par rapport au précédent zonage. Vos préoccupations sont légitimes. Je les partage et je vous confirme que le Gouvernement et l'ARS seront particulièrement vigilants.

sur demande des parents, à partir de 12 ans -s'établissait à 609 000 fin 2019. Un plan d'action a été défini pour résorber ces cartes surnuméraires. L'année 2019 avait déjà vu une réduction de l'excédent de cartes actives. Ainsi, 1,6 million de cartes ont été sorties du parc actif. À la fin du mois de mai, il restait 347 664 cartes surnuméraires, sur les 609 000 du début d'année. D'ici à fin octobre, ce nombre devrait encore baisser des deux tiers. Le dispositif Vitale est complexe, et de nombreuses actions ont été menées, depuis son origine, pour maîtriser le parc de cartes. Chaque régime mène sa propre gestion, en coordination avec les autres régimes et avec l'appui du GIE Sesam-Vitale. Au-delà de la gestion des cartes, il convient de rappeler que de nouveaux outils ont été mis en place pour sécuriser la gestion des droits. Outre les mises à jour périodiquement faites sur les cartes, l'assurance maladie a déployé un outil d'interrogation en temps réel des droits. point essentiel, car l'enjeu clé pour la maîtrise du risque réside bien dans la gestion des droits. En 2019, 240 400 professionnels de santé étaient utilisateurs et 213,2 millions de consultations des droits ont été faites. Vous évoquez une comparaison du nombre de cartes actives avec les chiffres de l'Insee qui dénombre la population présente sur le territoire. Nous comprenons tout à fait l'utilité de chercher à comparer les données. Toutefois, cette comparaison pose difficulté, car la logique de constitution et de gestion de ces bases est très sensiblement différente, comme les données recueillies. Le rapprochement entre les données de l'Insee, constituées sur une base partiellement statistique, et celles de l'assurance maladie, qui recense des personnes systématiquement identifiées et enregistrées à des fins de gestion, soulève plusieurs difficultés. Hors recensement, l'Insee opère chaque année une mesure par échantillonnage et procède à une extrapolation de l'évolution de la population. Une telle approche induit mécaniquement une première marge d'erreur.

C'est un bel effort, madame la ministre, mais la méthode que vous décriez est celle qui a été utilisée par l'Insee, la direction de la sécurité sociale, l'assurance retraite et l'assurance maladie dans un compte rendu du 5 septembre 2019 venu contrer les chiffres que nous avions trouvés. Pour nous contrer, la méthode est bonne

En plein confinement, l'effectif médical du service de pédopsychiatrie a conduit le centre hospitalier de Laval à fermer de manière provisoire le centre de consultation médico-psychologique (CMP) de Château-Gontier-sur-Mayenne. Cette décision a provoqué incompréhension et colère chez les familles d'enfants et d'adolescents qui ont besoin d'une prise en charge et d'un suivi régulier. Grâce à un mouvement solidaire local, à une mobilisation massive des élus locaux, des maires, des familles de patients et des professionnels de santé, les consultations au CMP de Château-Gontier vont pouvoir reprendre à la rentrée. C'est une première bonne nouvelle et une victoire. Cependant, les CMP d'Evron, d'Ernée et de Mayenne demandent aussi un engagement de votre part, madame la ministre, sur le maintien de leur activité en pédopsychiatrie. Ils ont besoin d'être rassurés. rassurés. Par le passé, les CMP décentralisés de Craon et de Pré-en-Pail ont fermé. Or ces établissements sont nécessaires, même vitaux, surtout en cette période de crise sanitaire post-confinement. Nous allons vers des situations graves si les enfants ne bénéficient pas de soins ou d'un suivi « psy » qui leur permettent de trouver une place dans notre monde. Pour leur bien-être et leur stabilité, il faut pérenniser l'accompagnement. Depuis cinq ans, les activités de pédopsychiatrie en Mayenne sont en difficulté, du fait de la diminution des effectifs médicaux, avec quatre équivalents temps plein (ETP) pourvus sur neuf théoriques pour cinq sites différents, dix structures et une file active d'environ 2 000 enfants par an. Cette situation en Mayenne est représentative d'un problème de démographie médicale majeur et pose, plus globalement, celui de la prise en charge de la santé mentale. Les grosses structures dont dépendent les CMP ferment des postes et des unités, ce qui fait baisser le nombre de médecins psychiatres. Ces derniers sont alors responsables de plusieurs pôles. Leur charge de travail et de responsabilité augmente en permanence. Ils finissent nécessairement par craquer. C'est surtout le cas dans les territoires ruraux.

et organiser l'offre de soins en santé mentale autour du patient et dans les territoires

L'intersecteur de pédopsychiatrie du centre hospitalier de Laval, qui couvre l'ensemble du département mayennais, a en effet vu son nombre de médecins pédopsychiatres décliner au fil des années. À la suite du départ de praticiens, seuls 3,2 ETP étaient pourvus en juin 2020, sur les 9,6 budgétés. Depuis le confinement, l'équipe du centre médico-psychologique a été regroupée au centre hospitalier de Laval, au pôle de psychiatrie, accessible par téléphone. À la sortie de la période de confinement, faute de disponibilité médicale suffisante, le centre hospitalier de Laval a décidé de fermer provisoirement le centre médico-psychologique de Château-Gontier à compter du 1 juin, avec reprise de certaines consultations à Laval, afin de garantir,, l'activité dans cette ville, dans l'attente de renforts médicaux. Cette situation montre la grande fragilité de la pédopsychiatrie mayennaise, qui doit faire face à des besoins croissants d'hospitalisation et de consultation, mais qui a su tisser des liens étroits avec tous ses partenaires. Devant cette situation particulièrement difficile, aggravée ces derniers mois, et qui menace la pérennité de la pédopsychiatrie lavalloise, l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a élaboré en juin, en lien étroit avec les acteurs concernés, un plan d'action portant sur la création d'un poste de praticien hospitalier partagé entre le Cesame, centre hospitalier spécialisé de Maine-et-Loire, et le centre hospitalier de Laval, sur une aide médicale ponctuelle d'urgence au CMP de Château-Gontier pour en permettre la réouverture,

on a pu obtenir qu'un médecin du CHU d'Angers se rende à partir de septembre prochain au centre médico-psychologique de Château-Gontier une fois par semaine, ce qui représente un doublement de la présence médicale par rapport à l'existant. ce médecin serait susceptible de prendre le poste partagé entre le Cesame et le centre hospitalier de Laval, une fois que ledit poste aura été publié. Outre son activité au CMP, il aura pour mission de créer un hôpital de jour sur ce secteur, et ainsi de renforcer l'offre. Une fois le recrutement de ce médecin entériné, nous pourrons annoncer une date de réouverture du CMP. La parole

Selon une enquête de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la Drees, parue le 14 février dernier, le désert médical n'en finit pas de s'étendre en France. Le nombre d'habitants vivant dans une zone sous-dotée en médecins généralistes est passé de 2,5 millions en 2015 à 3,8 millions en 2018, la Haute-Garonne n'échappe pas à cette réalité préoccupante. Les difficultés d'accès aux soins touchent de plus en plus de personnes ; les déserts médicaux s'étendent et vont continuer à croître, touchant les zones rurales comme certaines zones urbaines. À l'échelle nationale, 18 % de la population serait concernée, du fait de l'absence d'installation de jeunes médecins et de la désaffection pour l'installation libérale, sans oublier les aspirations à une réduction d'activité. Cette situation entraîne la mise en danger sanitaire de la population, notamment la plus fragile, et une précarité sanitaire qui se développe de façon alarmante. La mesure symbolique, contenue dans la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, de suppression du devrait certes certes permettre d'endiguer la pénurie de médecins, mais cette suppression ne sera effective qu'à la rentrée universitaire 2020. En outre, bien que l'objectif affiché d'augmenter d'environ 20 % le nombre de médecins formés soit louable, il faudra attendre une décennie pour que ses effets se fassent sentir. Une partie de la réponse pour faire face rapidement à la baisse de la démographie médicale et éviter une rupture d'équité territoriale réside dans la création de maisons de santé, regroupant soignants et professionnels de santé, proposant un exercice collectif et coordonné de la médecine.

pour faciliter leur déploiement ? Quelles solutions le ministère des solidarités et de la santé peut-il apporter pour pallier l'insuffisance des politiques publiques, conduisant à des inégalités territoriales en matière d'accès aux soins ? La parole

Cette situation est le résultat de plusieurs facteurs. Elle procède de mauvaises orientations- de 1991 à 2000, moins de 4 000 médecins ont été formés chaque année -et de problèmes d'anticipation : le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques n'ont pas été suffisamment pris en compte, l'évolution des pratiques des professionnels et des conditions d'exercice. Aujourd'hui, le département de la Haute-Garonne présente une densité médicale supérieure à la moyenne régionale et nationale, mais ce taux

partenarial à l'échelle du département et de la ville de Toulouse, plus spécifiquement en faveur des quartiers, avec l'appui de la ville de Toulouse et de son bailleur social. Les constats qui en découlent confortent la nécessité, pour l'ARS, de poursuivre et de renforcer l'accompagnement des structures d'exercice coordonné par diverses mesures.

; en réunissant tous les acteurs, je suis convaincue que nous trouverons des solutions adaptées à chacun des territoires ! La parole est à Mme

une femme sur cinq présente un lymphoedème du membre supérieur, et les lymphoedèmes du membre inférieur après cancer pelvien- cancer de la prostate chez l'homme ou cancer gynécologique chez la femme -touchent un patient sur quatre.

Ils sont donc susceptibles d'apparaître consécutivement à un traitement du cancer, et plus particulièrement à la suite du curage des ganglions sous l'aisselle, dans le cas du cancer du sein. L'incidence du lymphoedème secondaire post-cancer est insuffisamment connue, mais la Haute Autorité de santé, la HAS, estime qu'après cancer du sein celle-ci varierait selon le type de traitement le risque serait moins élevé chez les femmes qui subissent une biopsie des ganglions sentinelles que chez celles qui subissent un évidement des ganglions axillaires. Ainsi, la fréquence de survenue de cette pathologie est estimée actuellement entre 15 % et 28

Dans le cadre de la prise en charge au titre des affections de longue durée, ces actes sont remboursés à 100 % par l'assurance maladie. Quant au second objectif- l'amélioration de la qualité de vie des patients -, il passe par des conseils pratiques de vie au quotidien ainsi que par un bilan et un suivi d'activité physique, psychologique et diététique. À ce titre, le parcours de soins global après le traitement d'un cancer, créé par l'article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, dont les textes réglementaires sont en cours de finalisation, vise à améliorer la prise en charge des patients après le cancer sur l'ensemble du territoire en organisant la et la réalisation de bilans d'activité physique, psychologique et diététique, ainsi que des consultations de suivi psychologique et diététique. La parole

Le décret n° 2020-66 du 30 janvier dernier a instauré une prime « grand âge », versée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels relevant des grades d'aide-soignant dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, Cette prime mensuelle de 118 euros bruts, financée par l'assurance maladie, est destinée à reconnaître l'engagement des professionnels exerçant auprès des personnes âgées et à valoriser les compétences nécessaires à la prise en charge Le décret réserve cette prime aux agents des établissements sous statut public, excluant de fait les aides-soignants employés par les Ehpad privés à but non lucratif. Mon département, la Haute-Loire, compte 22 établissements de ce type, sur un total de 48 Ehpad. Cette mesure crée donc une forte inégalité entre les professionnels des Ehpad du secteur public et ceux du secteur privé à but non lucratif, alors même qu'ils exercent les mêmes missions, dans des conditions particulièrement difficiles. difficiles. Le recrutement de personnel dans les Ehpad n'est déjà pas aisé, et l'on constate une diminution des effectifs dans les instituts de formation : cette prime sélective ne fera qu'accentuer le déficit en personnel compétent dans les établissements du secteur privé. secteur privé. Le Gouvernement a-t-il l'intention de remédier à cette inégalité de traitement ? Envisage-t-il de généraliser la prime « grand âge » à l'ensemble des aides-soignants qui interviennent dans les Ehpad, quel que soit le statut de l'établissement qui les emploie ? La parole est à Mme la ministre déléguée.

qui justifient une meilleure reconnaissance financière des corps d'aides-soignants exerçant auprès des personnes âgées. Comme vous le constatez, le décret du 30 janvier dernier traduit cet objectif pour la fonction publique hospitalière. Dans le secteur privé, une telle revalorisation, si elle est encouragée, doit préalablement faire l'objet de négociations collectives entre les organisations représentatives des employeurs et les salariés. Les pouvoirs publics n'ont pas compétence pour se substituer aux partenaires sociaux dans ces négociations. L'État accompagne néanmoins la dynamique de celles-ci en fixant chaque année un taux de progression de la masse salariale du secteur social et médico-social privé à but non lucratif. Ainsi, pour l'année 2020, le Gouvernement a souhaité soutenir ce secteur en offrant aux acteurs les marges financières nécessaires pour instaurer une prime comparable à celle mise en place dans le secteur public. il a fixé un taux d'évolution de la masse salariale de 1,25 % pour l'ensemble des conventions collectives de la branche de l'action sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, et un taux différencié de 2,7 % pour la branche de l'aide à domicile. Cela représente un effort de plus de 310 millions d'euros en faveur des rémunérations du secteur social et médico-social, tous financements confondus. Le taux retenu ouvre aux acteurs du secteur privé non lucratif la possibilité de conclure des accords collectifs

La directive 2001/83/CE du Parlement européen, transposée à l'article R. 5121-138 du code de la santé publique, énumère limitativement les mentions devant figurer sur l'emballage extérieur des médicaments de manière à être plus facilement lisibles. Certaines mentions doivent également être indiquées en braille.

les fabricants. Je vous demande de bien vouloir me préciser la position du Gouvernement. Il convient d'obliger les entreprises destinataires de ces recommandations à les respecter, notamment en mentionnant sur les boîtes de médicaments des dates de péremption lisibles pour les personnes malvoyantes.

santé publique énumère ainsi les mentions devant obligatoirement figurer sur l'emballage extérieur du médicament, dont la date de péremption en clair, inscrite de manière à être facilement lisible, clairement compréhensible et indélébile.

orale solide. Elle insiste sur la nécessité de porter une attention particulière au choix de la police et de sa taille, afin de garantir la bonne lisibilité de l'ensemble des mentions et d'en faciliter la lecture, notamment par les personnes présentant des troubles de la vision et les sujets âgés.

deux chiffres ou au moins trois lettres pour le mois et quatre chiffres pour l'année. Enfin, la date de péremption doit également être mentionnée sur le conditionnement primaire des médicaments, c'est-à-dire le conditionnement avec lequel le médicament se trouve en contact direct. l'article R. 5121-138 du code de la santé publique prévoit que le nom et le dosage du médicament sont inscrits en braille sur le conditionnement extérieur ou, à défaut, sur le conditionnement primaire. sa décision du 7 mai 2008 prise en application de cette disposition, l'ANSM indique que, lorsqu'un espace suffisant est disponible, d'autres informations pertinentes peuvent être mentionnées en braille, dont la date de péremption. Le sujet de la lisibilité des informations disponibles est donc bien identifié. Une réflexion pourra et devra se poursuivre à ce titre avec le ministère chargé des personnes handicapées. La parole

Si nous demeurons le seul territoire français encore gravement touché, avec, aujourd'hui, plus de 6 700 personnes infectées, près de 150 patients hospitalisés, dont 34 en réanimation, et surtout 38 décès, ce n'est pas le fait d'un simple hasard c'est parce que les mesures prises pour anticiper et préparer la phase que connaît aujourd'hui la Guyane se sont révélées inadaptées et insuffisantes. Une fois de plus, il a fallu réagir dans l'urgence, avec les insuffisances de l'urgence de l'urgence ! Les Guyanais sont excédés. Ils ne supportent plus d'être discriminés, d'être considérés comme des citoyens de seconde zone en matière de santé, ce bien primordial, ce droit pour tous. Un mot d'ordre de grève générale est d'ailleurs lancé pour ce jour même.

et le redimensionnement des centres délocalisés de prévention et de soins de Saint-Georges-de-l'Oyapock et de Maripasoula en hôpitaux de proximité. Les élus, les syndicats, les collectifs citoyens et les organisations professionnelles tous ont relayé ces demandes en remettant une motion au Premier ministre lors de son récent déplacement en Guyane. Le ministre de la santé l'y accompagnait. Je sais qu'il doit présenter aujourd'hui même le second volet des mesures du Ségur de la santé, qui porte précisément sur l'organisation du système de santé. de santé. Vous l'aurez compris : la réponse du Gouvernement est vivement attendue

L'ensemble des mesures prises depuis plusieurs semaines jouent un rôle important dans la relative stabilisation de la situation épidémique en Guyane. Face à un important afflux de patients et au risque de saturation des capacités de prise en charge réanimatoire, une stratégie de réponse a été mise en place en Guyane. Elle repose sur quatre types de mesures et a pour objectif de maintenir la qualité des soins. Premièrement, l'envoi de matériels- respirateurs, appareils de monitorage, pousse-seringues électriques, etc. -et de consommables permettra d'armer des lits de réanimation, ou encore de répondre à un risque de pénurie de dispositifs médicaux nécessaires à la prise en charge des patients. Deuxièmement, l'envoi de médicaments nécessaires à la prise en charge de ces patients- hypnotiques, myorelaxants, etc. -permettra de répondre aux tensions d'approvisionnement. Troisièmement, le renforcement en professionnels de santé permettra d'atténuer et de mieux répartir la charge de travail qui pèse sur les professionnels, qui, vous l'avez rappelé, sont mis à rude épreuve, d'armer des lits supplémentaires et d'assurer les relèves. et enfin, l'évacuation sanitaire de patients permettra d'éviter l'engorgement de services risquant d'être saturés et d'accueillir de nouveaux patients. Depuis plusieurs semaines, les établissements de santé de Guyane prennent de nombreuses mesures pour renforcer les capacités hospitalières et faire face au covid-19, notamment dans les services de médecine et de réanimation : réorganisation des services, augmentation du temps de travail, déprogrammations, etc. Dans une logique de solidarité nationale, un appel à mobilisation a été lancé par le centre de crise sanitaire le 20 juin dernier, afin d'identifier des volontaires susceptibles de rejoindre les rangs de la réserve sanitaire pour être déployés en renfort sur le territoire guyanais. Le Gouvernement, sachez-le, est pleinement engagé, et nous ferons face à l'épidémie ensemble ! La parole

ces solutions figurent l'exercice coordonné sous toutes ses formes, dont on sait qu'il représente un fort levier d'attractivité, ou encore la télémédecine, qui permet d'abolir les distances- on en a vu l'efficacité pendant le confinement. Le déploiement de 400 postes de médecin généraliste en exercice partagé entre une structure hospitalière et une structure ambulatoire ou le salariat dans un centre de santé ou un établissement de santé fait effectivement partie des leviers supplémentaires annoncés dans le cadre de la stratégie Ma santé 2022 pour donner un nouvel élan à cette démarche, qui a permis d'engager assez vite une nouvelle dynamique. L'année 2019 a été celle du lancement de la mesure « 400 médecins ». En fin d'année, 110 postes avaient été pourvus en passe de l'être, grâce à l'engagement des ARS et de leurs partenaires pour proposer des offres attractives. Un nouveau bilan national sera fait très prochainement. D'ores et déjà, il s'avère que ce dispositif a permis de recruter vingt-trois médecins en Bourgogne-Franche-Comté, dont, plus

Nous avons fait le choix de la confiance aux acteurs pour innover et mettre en place des solutions adaptées aux contextes locaux, et nous avons pu observer que cette stratégie était la meilleure

territoriales. Madame la ministre, les dispositions de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN, étaient destinées à assouplir les restrictions imposées par la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

des équilibres biologiques. Parmi ces aménagements figurent, entre autres, les équipements légers et démontables nécessaires à la préservation et à la restauration de ces milieux, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, ou encore la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques. Ces dispositions sont certes bienvenues, mais elles ne laissent qu'une marge de manoeuvre étroite aux élus locaux qui souhaiteraient stimuler l'attractivité de leur commune littorale. À titre d'exemple, les équipements légers et démontables destinés à la restauration sur place ou à emporter ne répondent pas aux critères fixés par l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme. Les maires ne demandent rien d'autre que de pouvoir mettre en valeur les atouts de leur commune tout en préservant les caractéristiques patrimoniales et environnementales, ainsi que la biodiversité de leur littoral.

autorisés dans les espaces remarquables du littoral. Vous proposez d'étendre cette liste aux installations temporaires à vocation économique, pour répondre aux demandes des élus soucieux de l'attractivité de leur territoire. Depuis plus de trois ans, nous sommes mobilisés auprès des élus locaux pour renforcer le dynamisme de leurs territoires ; nous ne pouvons donc que vous rejoindre sur ce point. Je citerai le programme Action coeur de ville et les opérations de revitalisation des territoires. spécifiquement les communes littorales, la loi ÉLAN a également permis de faciliter les projets des communes, s'agissant notamment de traiter la problématique des « dents creuses » dans les zones littorales, qui faisait débat depuis des années.

La protection des espaces remarquables doit rester un objectif majeur de la loi Littoral. C'est pourquoi il n'est pas envisagé d'étendre les possibilités de dérogation au principe d'inconstructibilité qui régit ces espaces à des équipements qui seraient destinés à de la restauration sur place ou à emporter. De telles activités peuvent facilement générer des stationnements, voire, dans certains cas, des dépôts sauvages de déchets, dans des milieux à préserver particulièrement sensibles. Si, toutefois, certains projets respectant le caractère exceptionnel de ces espaces devaient se trouver empêchés, mes services sont disposés à étudier, en concertation avec la ministre de la transition écologique, ces difficultés et les exemples concrets que vous pourriez nous faire remonter.

Le Gouvernement a en effet souhaité définir une « nouvelle géographie prioritaire » de la ruralité pour accompagner l'évolution des dispositifs visant à réduire les inégalités territoriales. Le besoin de disposer d'une définition rénovée et positive des espaces ruraux est partagé, de même que celui d'une révision de certains zonages qui servent de base au soutien de l'État aux territoires, en particulier ruraux. Alors que le Parlement, notamment le Sénat, a produit de nombreux travaux sur ces sujets, à l'instar du récent rapport d'information sur les zones de revitalisation rurale fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et

Vous connaissez l'attachement des élus à leurs territoires, ainsi qu'aux dispositifs zonés, qui marquent le soutien de la Nation à leur égard. Aussi serait-il souhaitable que les décisions déterminantes pour l'évolution de ces zonages soient prises d'abord à un niveau politique, impliquant une large concertation des élus locaux et nationaux directement concernés. concernés. Pouvez-vous me confirmer que les parlementaires impliqués sur ce sujet seront effectivement associés à ces travaux et réflexions ? Monsieur le sénateur, vous nous interrogez, d'une part, sur l'articulation entre la définition de la ruralité et l'évolution du zonage prioritaire, et, d'autre part, sur l'association des élus, locaux et nationaux, à ces réformes. Conformément aux engagements pris dans le cadre de l'agenda rural, le Gouvernement a lancé conjointement deux exercices : un groupe de travail, piloté par l'Insee, est chargé de réfléchir à la définition statistique de la ruralité ; une mission inter-inspections, intégrant une large palette de compétences, doit proposer des pistes de réforme de la géographie prioritaire. Les travaux de l'Insee sont en cours. Le groupe de travail qu'il pilote implique plusieurs ministères et services de l'État, mais aussi des associations d'élus, afin d'aborder la question de la ruralité d'une manière aussi complète que possible. Ses membres ont réfléchi à l'emploi de nouvelles méthodes pour définir le phénomène rural autrement que comme une négation de l'urbain.

définitions ne sont pas seulement des catégories statistiques complexes, des catégories d'experts, mais produisent des effets dans la réalité. Elles cristallisent en effet une certaine vision de notre géographie et des territoires de notre pays. Nous veillerons donc à ce qu'un échange sur ce sujet puisse avoir lieu à un niveau politique. Le zonage prioritaire, qui est un zonage réglementaire, se distingue du zonage statistique ou d'étude. Les deux notions ont néanmoins vocation à être abordées simultanément, pour garantir la cohérence de l'action publique. Quant à la mission inter-inspections chargée de proposer des pistes d'évolution de la géographie prioritaire, elle vient de rendre son premier rapport. Constatant le caractère complexe, sédimenté, sédimenté, insuffisamment ciblé peut-être de notre géographie prioritaire, il a été conclu à la nécessité de la réformer. Le rapport de la mission inter-inspections, qui était chargée de nous proposer des scénarios, accorde une place de premier plan aux zones de revitalisation rurale, traite aussi des zones de restructuration de la défense, des « bassins urbains à dynamiser », ou encore des « bassins d'emploi à redynamiser ». Il se concentre spécifiquement sur l'efficacité des exonérations, fiscales ou sociales associées au classement dans ces zones prioritaires. Il esquisse trois grands scénarios d'évolution de ces exonérations : les rationaliser, déconcentrer leur attribution ou les supprimer et les transformer en crédits budgétaires gérés de manière décentralisée. Ces pistes se retrouvent d'ailleurs dans différents rapports parlementaires.

je souhaite attirer votre attention sur des dispositions qui appellent une clarification quant à leur application dans les départements d'Alsace et dans celui de la Moselle. Il s'agit, en premier lieu, deux dispositions contradictoires de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, dispositions relatives aux seuils à partir desquels les communes sont tenues de se doter d'un règlement intérieur. Avant cette loi, le droit local d'Alsace et de Moselle soumettait toutes les communes à l'obligation de se doter d'un règlement intérieur, mais l'article L. 2541-5 du code général des collectivités locales issu de la loi NOTRe a réservé cette obligation, en Alsace-Moselle, aux seules communes de 3 500 habitants et plus. Or l'article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales, également introduit par la loi NOTRe, a fixé le seuil à 1 000 habitants à compter de l'actuel renouvellement des conseils municipaux. De prime abord, cette dernière disposition apparaît applicable en Alsace-Moselle, car l'article cité n'y prévoit pas sa non-application. En attendant la nécessaire coordination législative entre ces deux dispositions, pouvez-vous me confirmer, madame le ministre, l'interprétation selon laquelle, en vertu de l'article L. 2541-5 du code général des collectivités territoriales,

En second lieu, j'aimerais que vous précisiez les modalités de convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal en Alsace-Moselle. En effet, la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique dispose que la convocation des conseillers municipaux se fait par voie dématérialisée,

est explicitement écartée par l'article L. 2541-1 du même code, et aucune disposition en la matière n'est prévue dans la partie du code consacrée au fonctionnement des communes de ces trois départements, à privilégier la convocation écrite traditionnelle. Il semble donc prudent de continuer, en Alsace-Moselle, d'envoyer les convocations par courrier.

Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur l'application de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux conseils municipaux des communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sachant que ces communes sont soumises à des règles de fonctionnement qui relèvent, pour certaines, du droit local. du droit local. Vous appelez notre attention, premièrement, sur les seuils à partir desquels les conseils municipaux sont tenus de se doter d'un règlement intérieur. Je ne rappellerai pas les modifications qui ont été apportées par la loi NOTRe- vous l'avez très bien fait dans votre question. L'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales prévoit l'obligation, à compter du renouvellement général de 2020, d'établir un règlement intérieur dans les six mois qui suivent l'installation du conseil municipal pour les communes de 1 000 habitants et plus. Cette obligation, comme vous l'avez comme vous l'avez souligné, ne s'imposait auparavant qu'aux communes de 3 500 habitants et plus. Pour ce qui concerne les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'article

imposait au conseil municipal de ces communes, quelle que soit leur taille, d'élaborer un règlement intérieur sans condition de délai. Même si aucune disposition du code général des collectivités territoriales n'écarte l'application de l'article L. 2121-8 aux communes de ces départements, il est en droit une règle fondamentale selon laquelle les lois spéciales dérogent aux lois générales. L'adoption d'un règlement intérieur n'est donc pas obligatoire pour les communes de moins de 3 500 habitants situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Vous appelez en outre mon attention sur l'application des modalités de convocation des conseils municipaux prévues à l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Cet article prévoit que la convocation au conseil municipal « est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Ce dispositif introduit par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique vise en effet à ce que l'envoi dématérialisé des convocations devienne la norme, et l'envoi par courrier l'exception. L'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales écartant explicitement l'application de cet article dans les communes des départements que nous avons cités, l'envoi par courrier des convocations au conseil municipal dans les communes de ces départements reste la norme. Il sera toujours possible, un prochain vecteur législatif, d'étendre cet envoi dématérialisé aux communes d'Alsace et de Moselle.

complexe, qui nécessite la recherche d'un équilibre constant entre la préservation justifiée de l'environnement et une urbanisation maîtrisée. Strictement encadrée, l'urbanisation dans les communes littorales a fait l'objet d'assouplissements, introduits par les dispositions de la loi du 23 novembre 2018, dite loi ÉLAN. Or l'interprétation stricte de ces dispositions, sans prise en compte des spécificités locales ou de la réalité économique, suscite de nombreuses incompréhensions chez les élus locaux concernés, ceux de la Seine-Maritime notamment. Deux sujets illustrent particulièrement ces difficultés. D'une part, il est impossible, pour les exploitants agricoles, de construire des locaux pour mettre en commun leurs productions et faire de la vente directe, au motif que cette activité n'est pas considérée comme « nécessaire » à l'activité principale

Or, dans le pays de Caux, les communes sont toutes constituées de nombreux hameaux, résultante du bocage normand. Ces hameaux sont d'ailleurs souvent beaucoup plus peuplés que le centre-bourg. Si Si l'urbanisation des communes littorales doit se faire dans le respect de notre patrimoine naturel, elle doit aussi prendre en compte les particularités locales des bourgs normands et l'évolution des pratiques agricoles.

Ma question est simple : comment mieux prendre en compte l'avis des élus locaux pour, sans déroger aux règles d'urbanisme, tenir compte des spécificités locales dans l'urbanisation des communes littorales ? La parole est à Mme la Madame la sénatrice, vous nous interrogez sur l'assouplissement de la loi Littoral pour les constructions agricoles. Pour répondre à la préoccupation de maintenir des activités agricoles en zone littorale, la loi Littoral a prévu une dérogation au principe Avant la loi ÉLAN, cette dérogation était soumise à une double contrainte : la construction ou l'installation devait être liée aux activités agricoles ou forestières et être incompatible avec le voisinage des zones habitées. Par ailleurs, les cultures marines n'entraient pas dans le champ d'application de cette dérogation, ce qui faisait obstacle au développement de cette activité. Devant ce constat et afin de répondre aux besoins des communes littorales de maintenir et de développer les activités réellement agricoles traditionnelles de leur territoire, nous avons, assoupli cette dérogation à deux titres : d'une part, en supprimant la condition selon laquelle les constructions en cause doivent être incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; d'autre part, en étendant le bénéfice de cette dérogation aux activités de culture marine, y compris dans les espaces proches du rivage. Il s'agit là d'assouplissements importants. En contrepartie, la loi ÉLAN a circonscrit le bénéfice de cette dérogation aux constructions ou installations réellement nécessaires, et non à celles qui sont simplement liées aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines. L'objectif est donc bien de favoriser les activités agricoles. Je

La Haute Assemblée, qui a particulièrement à coeur la défense des territoires, vient de se saisir d'une question d'importance pour ces derniers : celle de l'inclusion numérique, décrétée urgence nationale et voulue pour l'ensemble du pays. Le Sénat a constitué, le 13 mai dernier, une mission d'information, que j'ai l'honneur de présider, sur la lutte contre l'illectronisme, handicap invisible s'il en est et assez répandu en France à l'aube du XXI siècle.

Contre toute attente, les personnes âgées ne sont pas les seules concernées par cet illectronisme numérique. Toutes les classes d'âge, tous les milieux sociaux et, surtout, toutes les régions, urbaines comme rurales, sont concernés. Aussi, et parce que cette situation peut conduire nombre de Français à renoncer à leurs droits ou, pis encore, provoquer une exclusion sociale totalement inadmissible dans notre République, il convient de veiller à un juste équilibre dans les moyens mobilisés pour remédier à ce problème. Pour l'heure,

par tous les moyens à tous les Français, en particulier dans les zones rurales et les petites villes, est-il prévu, madame la ministre, que l'indulgence prévale quant à certaines démarches administratives obligatoires ?

sont loin d'être les seules concernées. Pour ces Français, la fracture est d'abord territoriale : 50 % des non-internautes résident dans des communes de moins de 20 000 habitants. Les niveaux d'études et de revenus sont également des facteurs déterminants d'inégalité. Le confinement a mis en lumière l'urgence à agir. En 2018, le Gouvernement a lancé une stratégie nationale pour un numérique inclusif, après une concertation avec les associations de collectivités territoriales et les grands opérateurs de service public. L'objectif est, premièrement, de consolider une offre de médiation numérique de proximité pour tous nos concitoyens, afin qu'ils puissent être accompagnés partout dans la réalisation de leurs démarches en ligne, et, deuxièmement, de permettre à chacun d'acquérir des compétences numériques de base utiles pour apprendre, échanger, trouver un nouveau travail. L'inclusion numérique est désormais une priorité gouvernementale, au nom de l'égalité des territoires et des citoyens. Deux dispositifs de la stratégie nationale pour un numérique inclusif concourent à apporter une solution au problème que vous soulevez. L'une des solutions qui ont émergé est le pass numérique, qui permet de financer des ateliers de médiation numérique contribuant à l'autonomie des publics éloignés

locales, pour favoriser le déploiement du pass numérique. Autre dispositif sur lequel le Gouvernement travaille depuis plusieurs mois : le service numérique Aidants connect. Cette solution a été développée au sein de l'incubateur des territoires de la nouvelle Agence nationale de la cohésion des territoires.

et d'ambitions. Les acteurs se sentent délaissés. Il faudrait des moyens appropriés pour former 13 à 14 millions de personnes au numérique. Cela ne se fait certes

territoriales. « Liberté, égalité, fraternité », telle est la devise de la République, une et indivisible. Or, dans la réalité, cet idéal reste verbal et s'évanouit lors de la répartition des dotations de l'État entre les villes et les campagnes. Ainsi, lorsqu'une commune de moins de 500 habitants bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement, ou DGF, calculée sur une base personnelle de 64,46 euros, une ville dont la population dépasse 200 000 habitants reçoit 128,93 euros par personne. Est-ce juste ? Cette différence, une véritable iniquité, est justifiée par vos services au nom des « charges de centralité » que doivent assumer les territoires plus peuplés, qui accueillent plus de services administratifs et commerciaux. Certes, les ruraux viennent chercher à la ville les services qu'ils n'ont pas, ou surtout plus, chez eux. Mais n'oublions pas que la loi du nombre aboutit pratiquement toujours à des coûts moyens d'investissement bien inférieurs en zone urbaine. Raccorder les 150 logements de l'immeuble d'un quartier au réseau d'assainissement d'une grande ville se révèle ainsi souvent moins onéreux qu'installer l'assainissement dans un hameau de 10 maisons. Cette problématique est d'ailleurs valable pour tous les réseaux : eau, électricité, téléphonie, fibre. Péréquation rime ainsi avec illusion en matière de soutien d'État aux territoires. Si les habitants des campagnes sont égaux devant l'impôt avec les urbains, ils ne le sont pas en termes de retour fiscal et d'offre de services. Les ruraux sont donc de bons contribuables, mais des citoyens de seconde zone. Au pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est-ce cohérent et acceptable ? En respectant la logique de votre administration, ne faudrait-il pas que l'impôt sur le revenu varie en fonction du lieu de résidence, puisque les habitants en milieu rural utilisent bien moins de services publics de proximité, faute de disponibilité ? Au nom de la solidarité nationale et de la justice territoriale, quand le Gouvernement révisera-t-il son algorithme, en apportant plus d'équité et de bon sens dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement ? La parole est à Mme la Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur la question de l'emploi d'un coefficient variant de 1 à 2 au sein de la dotation forfaitaire des communes. La question consiste à déterminer comment rendre compte, objectivement, des charges supportées par une commune dans son attribution de DGF. L'analyse économétrique conclut que les charges croissent avec la population. C'est ce qui explique pourquoi, au sein de la dotation forfaitaire, le gain d'un habitant conduit à un gain de dotation forfaitaire variant de 64 euros à 129 euros. Cet écart n'est pas apparu par hasard : il est fondé sur des travaux scientifiques conduits par des universitaires et plusieurs fois actualisés et confirmés. Le Gouvernement a publié un rapport détaillé sur la question l'année dernière, rappelant l'ensemble de ces analyses. Pour vous en convaincre davantage, monsieur le sénateur, je vais prendre deux exemples, qui, j'en suis certaine, vous parleront. Est-ce que l'on peut dire que, par habitant, que, par habitant, le niveau des charges contraintes supportées par la commune de Compiègne, soit un peu plus de 41 000 habitants, est le même que celui de communes voisines de 500 ou de 1 000 habitants Objectivement, la réponse est non, car il n'est tout simplement pas imaginable de ne pas prendre en compte les coûts, réels et objectifs, induits par la démographie dans la répartition des concours financiers de l'État. Par ailleurs, ce coefficient n'est qu'un critère parmi d'autres. Vous avez dû consulter la répartition de la DGF 2020 pour un certain nombre de communes de votre département de l'Oise. Vous avez dû constater que le niveau de la DGF totale ne varie pas du simple au double selon la population d'une commune, preuve que bien d'autres critères sont pris en compte et tendent à assurer, concrètement, une répartition équitable des concours de l'État. C'est le cas, par exemple, dans la dotation de solidarité rurale, Depuis 2017, le montant global de la DGF a été stabilisé, et la DSR a crû de 90 millions d'euros par an chaque année. ruraux, la DETR, a atteint depuis 2018 un niveau de plus de 1 milliard d'euros par an, soit un seuil jamais atteint par le passé. Enfin, nous avons lancé l'agenda rural, issu d'un travail de terrain, et ses nombreuses mesures en faveur de la ruralité et des habitants comme de ses élus. regard de ces éléments, vous voyez bien, monsieur le sénateur, que le Gouvernement ne se désintéresse pas du tout de la question de la ruralité. la réplique. Certes, le Gouvernement ne se désintéresse pas de la ruralité, j'en suis conscient. Néanmoins ce mode de calcul ne convient pas aux ruraux. Il existe une véritable ségrégation- je pèse mes mots qui s'illustre par ce chiffre qui va de 1 à 2. Ce n'est pas la DSR qui le comblera, même si les maires qui bénéficient d'un peu de DETR ou DSR en sont satisfaits.

des affaires étrangères. Monsieur le ministre, depuis l'annonce du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, nos concitoyens vivant au Royaume-Uni s'inquiètent de la situation fiscale, alors que la période de transition durera encore jusqu'au 31 décembre 2020. Lors de son audition au Sénat, Michel Barnier, chef de la Task Force pour la finalisation de l'accord, n'a rien caché des difficultés rencontrées pour arriver à un accord global avec le Royaume-Uni. Ma question a trait à la situation fiscale de nos compatriotes. Au début de l'année 2020, lors d'un déplacement en Écosse, nos compatriotes ont abordé les sujets qui les préoccupent au cours d'une réunion publique. La question des retraites pour ceux qui cotisent au Royaume-Uni a été prégnante. Ils craignent, en effet, que leurs trimestres ne soient plus reconnus suivant l'accord négocié. Il me paraît important, alors que les négociations sont en cours, d'attirer votre attention et celle de notre négociateur sur ce point. Quelle est votre mobilisation Au lendemain de la période de transition, les Français vivant au Royaume-Uni seront considérés comme résidant hors de l'espace économique européen. Seront-ils alors de nouveau assujettis au prélèvement de la contribution sociale généralisée, la CSG, et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS ? européenne, nos compatriotes ne bénéficient toujours pas de cette exonération malgré les nombreuses oppositions à la mise en place de cette mesure injuste. Je pense, notamment, à une pétition lancée à la fin de 2018 par les conseillers consulaires. Ces Français continuent d'être soumis à ces cotisations sans bénéficier d'aucune couverture sociale, de retraite ou de chômage. Il s'agit d'une discrimination et d'une véritable injustice au regard du principe d'égalité devant l'impôt. Il est donc urgent dès maintenant de penser l'après-Brexit. Pouvez-vous nous rassurer sur l'engagement du ministère sur ces deux points ? La parole

accompagner dans cette période chargée d'interrogations concernant le Brexit. L'accord de retrait entre l'Union européenne et le Royaume-Uni assure un maintien des droits acquis par les assurés ayant exercé leur mobilité avant la fin de la période de transition- le 31 décembre 2020 -, en ce qui concerne la totalisation des périodes pour la retraite et l'exportation des pensions de retraite dans les deux sens. C'est-à-dire que, en vertu de l'accord de retrait, ces droits acquis avant la fin de la période de transition ne pourront être remis en cause. En effet, les périodes d'activité des assurés français ayant travaillé au Royaume-Uni, réalisées avant la fin de la période de transition, seront prises en compte dans le cadre de l'ouverture et du calcul des droits à la retraite en France et au Royaume-Uni- même après la fin de la période de transition -, en application des règles de coordination de sécurité sociale des règlements européens qui continuent à s'appliquer. Les retraites britanniques et françaises continueront également à être versées à l'assuré selon le principe de « l'exportabilité », comme le prévoient les règles de coordination de sécurité sociale des règlements européens. Dès lors que l'assuré percevait déjà une pension avant la fin de la période de transition, celle-ci continuera à lui être versée dans son État de résidence. Ses soins de santé continueront à être pris en charge selon les règles de la coordination de sécurité sociale. Ainsi, et même après la fin de la période de transition, la France continuera à exporter les pensions des retraités d'un régime français, quel que soit leur lieu de résidence. S'agissant en revanche des personnes qui exercent leur mobilité entre le Royaume-Uni et la France après la période de transition, la situation demeure incertaine et dépendra de la négociation de la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Vous le savez, des négociations sont en cours pour parvenir à un accord régissant cette relation après le 31 décembre 2020. Le mandat de négociation de l'Union européenne sur la relation future prévoit bien- c'est -que « le partenariat envisagé devrait traiter la question de la coordination en matière de sécurité sociale ». Les dispositions qui seront adoptées et les droits qui en découleront dépendront donc du résultat des négociations. Nous devons nous préparer à la possibilité d'un- il est important de l'avoir en tête -à l'issue de la période de transition. Dans cette hypothèse, le Gouvernement sera habilité à prendre par ordonnances des mesures nécessaires à la préservation de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou exerçant une activité, mais ces mesures seront soumises à une stricte réciprocité ; elles ne pourront donc être mises en oeuvre que si les autorités britanniques assurent les mêmes droits aux ressortissants français au Royaume-Uni.

de l'Europe et des affaires étrangères. Le département de la Savoie est très dépendant du tourisme, hiver comme été. Les citoyens britanniques représentent une large part des touristes de nos stations ; de même pour les salariés de même provenance qui accompagnent ces voyageurs et renforcent les équipes en place pour un accueil adéquat. Les tour-opérateurs qui organisent ces voyages en France sont aujourd'hui inquiets, car à l'issue de la période transitoire le 31 décembre 2020 le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Les contours de cette sortie restent encore flous. Deux cas de figure se présentent à eux : soit les saisonniers britanniques sont recrutés par une entité française avec un contrat de droit français avant le 3 décembre 2020, et ils ne savent pas si après cette date le contrat, même antérieur, sera toujours valable et si les saisonniers auront besoin d'une autorisation de travail pour terminer la saison sur le territoire national soit, dans l'hypothèse où la qualité de travailleur détaché est validée, même postérieurement au 31 décembre 2020 entre nos deux pays, ils ne savent pas non plus s'il sera nécessaire d'obtenir une autorisation de travail pour terminer ce contrat. Par ailleurs, monsieur le ministre, même si ce point ne vous concerne pas directement, je souhaite profiter de cette question orale pour alerter le Gouvernement sur le fait qu'Eurostar a annoncé que ses trains ne rejoindraient plus les destinations de montagnes du département comme ils le faisaient de Londres vers Moûtiers, Aime-la-Plagne ou Bourg-Saint-Maurice pour déverser les flots de touristes britanniques au pied des stations de montagne les plus renommées au monde. Une telle décision aurait un impact considérable non seulement sur le tourisme, mais aussi sur le bilan carbone de ces déplacements, la seule possibilité restant alors l'acheminement par avion jusqu'à l'aéroport de Chambéry-Voglans, puis par bus. par bus. Ces contraintes constituent des freins à l'essor économique, voire à la reprise économique et à l'emploi dans les territoires de montagne et de notre pays tout entier. En effet, elles risquent de décourager de nombreux touristes, des tour-opérateurs et des travailleurs britanniques. Aussi, j'aimerais, monsieur le ministre, que le Gouvernement apporte par ses réponses une meilleure visibilité à l'ensemble des entreprises de l'économie touristique de montagne, à leurs saisonniers et aux élus. La parole

de la clientèle britannique pour notre industrie touristique, en particulier en Savoie, et du rôle des saisonniers britanniques pour l'accueil de ces touristes. C'est pourquoi nous sommes très attentifs aux conséquences du retrait du Royaume-Uni

j'ai constaté comme vous qu'Eurostar avait décidé de ne pas assurer le service à destination des Alpes cet hiver. Il faut rappeler que la crise du covid-19 a eu un impact particulièrement fort sur Eurostar du fait de sa nature d'opérateur transfrontalier. L'incertitude liée à l'évolution de la situation sanitaire ne leur permet pas permet pas non plus d'envisager un retour rapide de la demande. C'est dans ce contexte difficile qu'Eurostar a prévu un plan d'économies drastique, ainsi qu'une réduction de sa flotte, donc de son plan de transport, en se concentrant sur les principaux itinéraires.

S'agissant des conditions de séjour des touristes britanniques en France, l'accord de retrait, entré en vigueur le 1 février dernier, garantit les droits liés au séjour des ressortissants britanniques. Pendant la période de transition, qui devrait en principe s'achever le 31 décembre, le voyageur britannique doit être muni d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité. Aucun visa n'est nécessaire. S'agissant des conditions d'emploi des travailleurs saisonniers britanniques, pendant la période de transition, la réglementation européenne relative au détachement des travailleurs reste applicable. La possibilité de poursuivre les détachements en cours à l'issue de la période de transition dépendra de la conclusion d'un nouvel accord portant sur la relation future, faute de quoi ils prendront fin au 31 décembre 2020. En l'absence d'accord à l'issue de la période de transition, nous serons tenus d'appliquer les dispositions de droit commun régissant les conditions dans lesquelles des ressortissants de pays tiers peuvent entrer ou séjourner dans l'Union européenne en tant que travailleurs saisonniers. C'est la directive de 2014 relative aux ressortissants britanniques. Comme vous, je regrette cette incertitude, mais elle n'est que le reflet de celle, plus générale, pesant sur nos relations futures avec le Royaume-Uni. Il faut continuer de se préparer aux conséquences d'un éventuel à la

Merci des outre-mer. La crise sanitaire et économique que nous traversons participe, partout en France, à l'augmentation des prix à la consommation. C'est vrai dans l'Hexagone. C'est particulièrement visible dans les outre-mer. Cette situation est évidemment difficile à accepter pour nos compatriotes ultramarins. Tout d'abord, parce que la pauvreté et le chômage y sont plus élevés qu'ailleurs. En Guadeloupe, pour ne prendre que cet exemple, un tiers de la population- c'est-à-dire près de 135 000 personnes - vit au-dessous du seuil de pauvreté. Ensuite, parce que les écarts de prix constatés avec l'Hexagone sont particulièrement importants, en raison de l'éloignement, bien sûr, et des frais de transport que la distance provoque, en raison aussi d'un manque criant de concurrence dans le secteur de la grande distribution. Le code de commerce autorise pourtant le Gouvernement, en Guadeloupe et dans certains territoires d'outre-mer, à réglementer, voire à encadrer, le prix de vente de produits de première nécessité et de consommation courante. L'article L. 410-2 du même code autorise d'ailleurs le Gouvernement à arrêter « des mesures temporaires motivées par une situation de crise, par des circonstances exceptionnelles ou par une calamité publique ». Ma question, monsieur le ministre, est la suivante : quelles mesures entendez-vous prendre dans les outre-mer pour contenir rapidement une hausse des prix aux effets potentiellement dévastateurs ?

en 2017. Parmi les mesures en place, on peut souligner les accords de modération des prix, ou « bouclier qualité-prix », renforcé en 2020 par la création de trois catégories de produits assorties chacune d'un prix maximal, notamment pour les produits alimentaires, les produits d'hygiène et les produits pour la petite enfance. On peut également souligner la création des observatoires des prix, des marges et des revenus, et des revenus, dont les moyens ont été doublés en 2019 à 600 000 euros et reconduits pour 2020. Des référents « vie chère » ont également été nommés au sein des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), pour assister les observatoires

a été mise entre parenthèses pendant la crise sanitaire. Plusieurs enquêtes d'observation des prix des fruits et légumes ont été menées par les Direccte sur les marchés de gros et de détail pendant le confinement. Aucune tension inflationniste particulière n'a été constatée. Différents décrets ont été pris, afin de réglementer les prix des masques et les gels hydroalcooliques en métropole, dans les départements-régions d'outre-mer, les DROM, les trois Saintes et à Wallis-et-Futuna. De plus, les produits nécessaires à la lutte contre la covid-19 ont fait l'objet d'une exonération d'octroi de mer sanitaire. sanitaire. Enfin, l'enjeu de la lutte contre la vie chère en outre-mer aura toute sa place dans le cadre du plan de relance économique, cela va sans dire. En effet, si le renforcement des mesures de contrôle doit être poursuivi, il est également essentiel d'accompagner la concurrence dans ces marchés et l'arrivée ou le développement de nouveaux acteurs économiques. Le plan de relance comprendra différentes mesures de financement des entreprises. Je veillerai personnellement, avec le ministre de l'économie, des finances et de la relance, à ce qu'elles renforcent la production locale et la concurrence, qui, parce qu'elles sont parfois défaillantes dans ces territoires, conduisent à des prix

à 12,5 % plus élevés dans les départements d'outre-mer, et supérieurs de 19 % à 38 % pour les seuls produits alimentaires. L'urgence est donc double et l'action du Gouvernement indispensable, qu'il s'agisse de réguler les prix à la consommation des produits de première nécessité et de consommation courante ou de stimuler une concurrence en matière d'importations et de distribution des produits de grande consommation,

la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats de Mayotte. L'article 2 du décret du 26 novembre 1996 prévoit qu'« une affectation à Mayotte ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation de deux ans hors de cette collectivité ou d'un territoire d'outre-mer ». L'article 4 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires est venu abroger ce décret de 1996. Ledit décret prévoit néanmoins,

-fait obstacle à l'application des dispositions du présent décret, pendant toute la durée de leur affectation dans le département de Mayotte durant laquelle ils sont régis par les dispositions du décret du 26 novembre 1996 Cependant, ces dispositions continuent en pratique à être opposées à certains fonctionnaires affectés après la date d'entrée en vigueur du décret dans ce département. Je vous demande donc de préciser l'interprétation des dispositions relatives à la mobilité des fonctionnaires de l'État à Mayotte.

1996, qui, d'une part, limitaient les durées d'affectation dans ces territoires à deux ans, avec une possibilité de renouvellement, et, d'autre part, excluaient la possibilité d'une mutation d'un territoire à l'autre au terme de cette période, en considérant que ces quatre territoires avaient des régimes équivalents. La départementalisation de Mayotte, vous l'avez rappelé, a été l'occasion, avec la parution d'un nouveau décret du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés, pour les magistrats et fonctionnaires de revenir en partie sur ces contraintes. Ainsi, les affectations à Mayotte ne sont plus limitées dans le temps et sont donc désormais régies par le droit commun. Toutefois, la disposition sur la possibilité d'une mutation directe entre Mayotte et les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna n'a pas été supprimée au même moment. Cette disposition avait un sens quand les quatre territoires obéissaient à des régimes équivalents et qu'il convenait de les considérer, notamment pour les modalités d'affectation, comme relevant d'un même périmètre. ce n'est plus cas aujourd'hui, si bien que cette restriction à la mobilité depuis Mayotte vers la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, ne paraît aujourd'hui pas conforme à l'esprit du nouveau statut de Mayotte et peut être vue comme une rupture d'égalité. Afin d'y remédier, des instructions seront transmises dans les plus brefs délais aux ministères pour permettre sans attendre aux agents qui le souhaitent d'effectuer leur mobilité. Il est par ailleurs également envisagé de modifier dès que possible, l'article 2 du décret

Les dépôts sauvages d'ordure empoisonnent littéralement nos communes. Par le fait de quelques-uns, des paysages sont défigurés. Le confinement a malheureusement aggravé cette situation. Certes, il s'agit d'un problème ancien, qui se fonde avant tout sur l'incivisme de quelques personnes, mais ses implications sont lourdes de conséquences : entre 340 et 420 millions d'euros pour

jetés normalement. La charge de la verbalisation et de l'identification des dépôts incombe aux maires des communes concernées, mais, dans de nombreux cas, ceux-ci se disent dépassés par ces incivilités. Qui plus est, la question des déchets est souvent une compétence de l'agglomération, ce qui éloigne d'autant le problème de la solution. Si les cadres légaux relatifs aux peines à appliquer sont clairs, de nombreux élus témoignent de leurs difficultés à les faire appliquer, car ils sont le plus souvent seuls face aux contrevenants quand ils sont identifiés. Le drame de Signes, commune dont le maire, Jean-Mathieu Michel, a été a été tué alors qu'il s'apprêtait à verbaliser le responsable d'un dépôt sauvage, est dans tous les esprits. Madame la ministre, il est très urgent de trouver une solution à ces problèmes. problèmes. J'aimerais connaître les moyens effectifs que l'État met à la disposition de tous les maires, en premier lieu en termes de prévention, mais également en termes d'appui à l'investigation et à l'application des textes réglementaires. La parole

qui m'a chargée de vous répondre. Le Gouvernement a fait de la lutte contre les dépôts sauvages l'une de ses priorités. La loi anti-gaspillage de février 2020 a permis de nombreuses avancées. Tout d'abord, pour agir à la source, une filière à responsabilité élargie du producteur sera créée le 1 janvier 2022 pour les déchets du bâtiment, ce qui permettra de constituer un maillage efficace en points de reprise et une reprise gratuite pour les déchets triés. Ensuite, pour financer le nettoyage des dépôts sauvages, les filières concernées prendront en charge une partie des coûts. Le projet de décret d'application de cette mesure fait actuellement l'objet d'une consultation du public. De plus, les amendes administratives payées par les auteurs de dépôts sauvages sont perçues par les collectivités, apportant ainsi un complément budgétaire en contrepartie de leur mobilisation contre ces dépôts. Enfin, la loi renforce les sanctions pour les rendre dissuasives. Elle sera complétée par un renforcement de la contravention pénale sanctionnant les petits dépôts sauvages, qui passera de la troisième à la quatrième classe. Le projet de décret concerné a été discuté avec les parties prenantes dans le courant du mois de juin dernier et sera publié à la fin de l'été. La loi prévoit également plusieurs mesures pour faciliter le travail au quotidien des élus. L'accès au système d'immatriculation des véhicules et l'utilisation de la vidéosurveillance facilitent l'identification et la sanction de l'auteur du dépôt sauvage. Les moyens humains et financiers peuvent être mutualisés au niveau des groupements de collectivités. Enfin, les agents de surveillance de la voie publique peuvent dès à présent sanctionner les dépôts sauvages. Un décret, qui sera présenté prochainement au Conseil national d'évaluation des normes, le CNEN, permettra d'habiliter d'autres agents choisis par les collectivités. Le groupe de travail sur le sujet, lancé en 2018 et rassemblant l'administration, des élus locaux, des parlementaires et les autres parties prenantes, poursuit ses travaux pour continuer à identifier de nouvelles actions, comme la formation des agents des collectivités locales. La parole

pour savoir si ceux-ci avaient déjà été victimes d'agressions dans le cadre de leur action. Quelque 92 % des maires ayant répondu ont déclaré avoir déjà été pris à partie dans le cadre de leur mandat 45 % d'entre eux ont été victimes d'actes de malveillance en tentant de rétablir l'ordre. Il faut donc aujourd'hui prendre de véritables mesures et aider

Très éloigné du projet d'amélioration des mobilités qu'appelle l'intense trafic de cette gare, ce projet est purement financier et anti-écologique. La SNCF et, surtout, son associé le groupe Auchan, qui détient 66 % du projet sa filiale immobilière Ceetrus, cherchent à capter commercialement 200 millions d'usagers annuels en transformant en centre commercial plus de 20 000 mètres carrés de la nouvelle gare au détriment des usagers. Ce projet sera un gâchis du même acabit que l'inutile et nuisible Charles-de-Gaulle Express, allant à l'encontre du rééquilibrage nécessaire des activités dans Paris et dans l'espace de la métropole du Grand Paris. Les commissaires enquêteurs qui ont approuvé le projet reconnaissent eux-mêmes que l'insertion urbaine et le trafic banlieue- rien que cela ! -sont maltraités par le projet. De nombreux acteurs et élus- le Comité des habitants Gare du Nord-La Chapelle, la mairie de Paris, un collectif de 19 architectes et urbanistes de renom -estiment négatives les conséquences du projet, pour les usagers comme pour les riverains. D'autres choix sont appelés, et sont possibles, pour faire de la gare du Nord un espace civilisé de mouvement et de rencontres. La Ville de Paris a annoncé qu'elle allait engager des recours contre ce projet d'un autre temps, en contradiction avec les exigences de la transition écologique. Madame la ministre, le Gouvernement compte-t-il retirer ce projet pour ouvrir la voie à une remise à plat, ou va-t-il s'entêter ?

s'est tenue entre le 20 novembre 2019 et le 8 janvier 2020. Au terme de cette enquête, la commission d'enquête a rendu un avis favorable le 25 février 2020. Dans les réponses aux questions de la commission d'enquête, les porteurs de projet ont pris 13 engagements visant à assurer la meilleure intégration possible de la gare rénovée dans le quartier, avec notamment la création d'un important parking à vélos, le lancement d'études pour améliorer l'accès à la gare par le nord et la prise en la prise en compte du réaménagement du parking souterrain pour pouvoir libérer le parvis de la gare des dépose-minute, tout cela afin de rendre ce projet écologiquement exemplaire. Conformément aux recommandations de la commission d'enquête publique, les discussions se sont encore poursuivies ces dernières semaines avec la Ville de Paris, sous l'égide du préfet de la région d'Île-de-France. Dans la dernière version du projet, les surfaces des activités commerciales ne constituent nullement une entrave au fonctionnement de la gare. Leur proportion se situe strictement dans la moyenne des autres gares parisiennes réaménagées récemment. les commerces contribuent au financement des investissements dans l'ensemble de la gare, au bénéfice du confort des voyageurs. Prenant acte de l'avis favorable de la commission d'enquête et des engagements de la société d'économie mixte à la société Gare du Nord 2024 le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sur le projet de transformation de la gare du Nord. La délivrance de ce permis de construire est une pour l'aménagement de la gare du Nord. Elle permettra à celle-ci de se situer au niveau des autres grandes gares européennes en termes tant d'équipements, d'accessibilité et d'intermodalité que de capacité. Le lancement des travaux aura donc lieu. Nous veillerons à ce que les riverains, les usagers, les commerçants et les élus restent étroitement associés au déroulement de ceux-ci, notamment au sein du comité des parties prenantes qui sera mis en place pour limiter les nuisances et les désagréments.

par le groupe Auchan, qui n'a rien, à ma connaissance, d'un groupe ferroviaire ... Il s'agit donc à l'évidence d'un projet dominé par les exigences commerciales. Contrairement à ce que vous avez

réélus, sont clairs à ce sujet. Si vous vous entêtez, vous allez voir surgir une contestation grandissante contre ce projet au coeur de Paris, alors que les urgences en matière de transport ferroviaire et de rénovation de la gare sont, elles, extrêmement importantes- mais ce n'est pas ce projet qui permettra

L'article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression intégrale de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour 80 % des ménages et une suppression progressive pour les 20 % restants. À compter de janvier 2023, tous les contribuables anciennement assujettis à la taxe d'habitation au titre de leur résidence principale ne seront plus concernés par cette taxe. Je vous rappelle que, actuellement, le troisième alinéa de l'article 1530 du code général des impôts prévoit une répartition de cette taxe entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, En réponse à une question écrite posée par notre collègue Jean-Raymond Hugonet, le Gouvernement a indiqué le 14 mars 2019 prévoir des aménagements du calcul de la taxe Gemapi, notamment dans le cadre de la refonte de la fiscalité locale et du financement des collectivités locales. Nous apprenons, par le biais d'une note d'information du ministère de la cohésion des territoires et des collectivités territoriales du 28 février 2020, qu'il est prévu que, à compter de 2023, la taxe Gemapi sera répartie entre les redevables des taxes foncières, des taxes foncières, de la CFE et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, au prorata des recettes que chacune de ces taxes aura procurées l'année précédente. Cela signifie donc un alourdissement fiscal important de cette taxe vers les propriétaires et les entreprises. Ce transfert semble favorable aux locataires et défavorable aux propriétaires bailleurs, puisque l'ensemble des locataires de leurs résidences principales se verront exonérés de cette taxe. Jusqu'alors, seuls les organismes HLM et leurs occupants en étaient exclus. À cet alourdissement de la fiscalité pour les propriétaires bailleurs viendra s'ajouter la mise en oeuvre du plafonnement des loyers dans les zones tendues. Aussi, un propriétaire appliquant le montant plafond subira obligatoirement une diminution de ses revenus locatifs. Madame la ministre, quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre afin de limiter les conséquences financières

Comme vous le savez, la taxe Gemapi est une taxe facultative, additionnelle aux quatre taxes directes locales, perçue exclusivement au profit des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, à fiscalité propre qui exercent cette compétence Le produit de la taxe est arrêté annuellement par l'organe délibérant de l'EPCI qui l'a instituée et votée, dans la limite d'un plafond de 40 euros par habitant résidant sur le territoire de l'EPCI. Il ne peut dépasser le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence Gemapi. Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, la CFE, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente sur le territoire de l'EPCI à fiscalité propre qui l'instaure, aux communes membres de ce dernier et aux syndicats dont elles sont membres. La suppression totale et définitive, par étapes, de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale conduit à une nouvelle répartition de la taxe Gemapi, qui portera à terme sur les redevables des taxes foncières, de la taxe d'habitation afférente aux résidences secondaires, ainsi qu'aux autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, et de la CFE. Dans la mesure où la taxe Gemapi concourt, à titre principal, à la protection des propriétés bâties et non bâties, il n'apparaît pas illogique que cette taxe se concentre davantage sur les impôts des propriétaires. En outre, l'institution de la taxe demeure facultative, l'organe délibérant pouvant décider de financer la compétence Gemapi par d'autres ressources, telles que les recettes non affectées du budget principal, par exemple. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de mesure spécifique relative à cette compensation.

Mme la ministre du travail sur les initiatives publiques locales destinées à faciliter la mise en oeuvre de la formation professionnelle des jeunes. En milieu rural éloigné des centres urbains, où se concentre l'essentiel des établissements d'enseignement professionnel, la faible mobilité des personnes concernées liée à la rareté de l'offre de transports collectifs et au coût d'obtention du permis de conduire, sans compter celui de l'acquisition d'un véhicule, aggrave la situation. Les quelques centres de formation des apprentis ou les lycées professionnels présents dans la ruralité manquent d'internats et de dessertes de transports et doivent redoubler d'ingéniosité pour faciliter l'accès à leur établissement. En complément des aides à la personne- transports, hébergement et restauration -consenties par les conseils régionaux, les communes ou les intercommunalités interviennent souvent à leurs frais pour organiser les liaisons avec les gares routières et ferroviaires les plus proches, ou trouver des solutions d'hébergement de proximité. proximité. Ces interventions, « facultatives », mais animées de la volonté d'appuyer les établissements et d'offrir davantage de chances aux jeunes ruraux, mériteraient d'être évaluées et soutenues financièrement par l'État. Le Gouvernement envisage-t-il de prendre en compte l'intérêt de ces initiatives publiques locales pour la mise en formation des jeunes et de les rendre éligibles à un soutien financier ? La parole Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice Nadia Sollogoub, je vous remercie de votre question. Vous avez tout à fait raison, la question de la formation est essentielle lorsque l'on parle de l'insertion des jeunes. Vous l'avez rappelé, les jeunes sans qualification ont le plus fort taux de chômage de la population française. Cependant, le Gouvernement n'a pas attendu la crise pour agir en faveur de leur formation. Je pense tout d'abord au Plan d'investissement dans les compétences, 13,8 milliards d'euros sur le quinquennat pour former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi, ce n'est pas rien ! Je pense aussi à l'apprentissage, qui a été réformé en 2018, de le rendre plus simple et lui redonner l'attractivité qu'il mérite pour les jeunes et les entreprises. En 2019, nous avons constaté une augmentation sans précédent du nombre de contrats d'apprentissage, avec une croissance à deux chiffres, notamment dans le secteur du BTP

La mise en place du service public de l'insertion et de l'emploi, le SPIE, est l'un de mes objectifs prioritaires. Je vais d'ailleurs me rendre prochainement dans les 14 départements expérimentateurs. Ma méthode est celle d'une élue locale : aller sur le terrain et prendre en compte les spécificités de chaque territoire. C'est notamment dans ce cadre que des réponses seront apportées aux problématiques du logement et de la mobilité des jeunes que vous mentionnez. mentionnez. Enfin, face à la crise, le Gouvernement a annoncé un plan pour l'emploi des jeunes. Il comportera un soutien à l'embauche à hauteur de 4 000 euros pour un contrat long ; un plan de relance de l'apprentissage, avec une prime de 5 000 euros pour les moins de 18 ans et de 8 000 euros pour les plus de 18 ans ; 300 000 contrats et parcours d'insertion pour les plus éloignés de l'emploi ; enfin, 100 000 services civiques jeunes de s'engager dans des missions utiles à la société. Madame la sénatrice, le Gouvernement n'a qu'un objectif : pas un jeune sans solution en septembre ! Nous y veillerons, nous nous y engageons. La situation l'exige et nous serons à la hauteur.

Les aides financières sont une chose ... Mais que faire d'un bon de transport lorsqu'il n'y a pas de transport public ? Pour cette raison, certains maires- j'ai en tête l'exemple de la commune de Varzy, dans la Nièvre -veillent à mettre en place une navette communale pour emmener les jeunes à la gare le vendredi soir et les ramener le lundi matin, ce qui représente plusieurs dizaines de kilomètres et, bien entendu, une charge financière. D'autres recensent les chambres chez l'habitant ou ont des projets d'aménagement de bâtiments communaux pour y faire des studios destinés spécifiquement aux apprentis. Néanmoins, ces élus ne sont pas soutenus financièrement pour ces projets. Ils mettent pourtant en place des services indispensables

Mme la ministre de la culture. Madame la ministre, le marché du livre d'occasion, particulièrement celui de la bande dessinée, a pris une importance considérable ces dernières années. Le prix d'occasion des livres est régulièrement, sinon systématiquement, affiché à côté de leur prix neuf, ce qui est fortement incitatif pour les clients. Ce nouveau marché marché de l'occasion enrichit tous les acteurs, à l'exception notable des auteurs et des éditeurs, lesquels sont pourtant les premiers concernés. Il ne s'agit plus d'un phénomène lié aux fêtes de fin d'année, à l'occasion desquelles une colossale quantité d'ouvrages à peine reçus en cadeaux sont sitôt proposés à la vente sur internet, des plateformes détenues par des géants mondiaux. Cette pratique pose des problèmes économiques et juridiques de grande ampleur. Hier marginal, le marché de l'occasion représente aujourd'hui plus de 42 % des ventes de livres. Ses acteurs, parmi lesquels Amazon, PriceMinister, la FNAC ou eBay, touchent des commissions sur chaque vente et sont soumis pour partie à la taxe En revanche, ceux qui ont créé et édité les livres vendus ne perçoivent aucun bénéfice de cette exploitation et voient même leur chiffre d'affaires amputé de recettes non négligeables. En effet, une l'étude qualitative menée par l'institut GfK à l'occasion des Rencontres nationales de la librairie, en 2017, indiquait que 16 % des acheteurs de bandes dessinées et 25 % des acheteurs de livres, tous genres confondus, déclaraient acheter des ouvrages d'occasion. Ramené aux 4 milliards de chiffre d'affaires de l'édition, cela représente un manque à gagner de 800 millions à 1 milliard d'euros. Dans le cas de la vente d'occasion, seuls le libraire, le site, le vendeur et, dans une moindre mesure, l'État touchent un pourcentage. Face au développement de la vente d'occasion, les créateurs, les auteurs et les éditeurs sont donc fortement pénalisés. Les premiers sont en effet privés d'une part non négligeable de leurs droits d'auteur et les seconds voient baisser significativement leurs ventes moyennes, ce qui rend leurs coûts de création de plus en plus difficiles à amortir et met en péril financier l'ensemble du secteur de l'édition. C'est pourquoi il semble nécessaire de réglementer la vente de livres d'occasion. La majorité de ces ventes se faisant sur les grandes enseignes de vente en ligne, nous pourrions imaginer obtenir de leur part un déclaratif de ces ventes et, à travers un organisme collecteur, obtenir un reversement destiné aux auteurs et aux éditeurs. Face à l'accroissement de la vente d'occasion, les créateurs, les auteurs et les éditeurs, vous le voyez, sont fortement pénalisés. Aussi, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer quelles sont les pistes qui peuvent être mises en oeuvre pour réglementer cette vente du livre d'occasion. La parole est à Mme la ministre. Monsieur

cela me mobilisera au cours des mois à venir. Vous me pardonnerez de ne pas être complètement d'accord avec le diagnostic que vous avez posé sur le marché du livre d'occasion. Selon les données du ministère de la culture relatives aux évolutions des pratiques d'achat, si d'achat, si ce dernier est en progression, il reste limité, puisqu'il représente moins de 8 % des sommes dépensées par les ménages pour leurs achats de livres en 2019. En outre, si les opérateurs que vous citez occupent une place importante sur ce marché, un achat de livre d'occasion sur deux s'effectue directement de particulier à particulier, notamment dans les bourses aux livres scolaires, les marchés ou les brocantes, que je sais nombreuses dans votre département du Nord. Les auteurs ne sont pas privés d'une partie de leurs droits d'auteur, dans la mesure où ils ont exercé leur droit exclusif de commercialiser les exemplaires de leurs oeuvres, l'exercice de ce droit de distribution entraînant son épuisement. Au-delà, la création d'un droit de suite des auteurs de livres n'est pas autorisée par les textes internationaux et européens. Vous évoquez aussi l'idée d'un reversement de la part des grandes enseignes de la vente en ligne.

suite des sollicitations de Bergerault Percussions, cet EPCI a finalement modifié son appel d'offres en incluant de nouvelles marques, mais toujours sans citer les principales marques françaises. À l'heure où nous souhaitons favoriser et recentrer la production artisanale et industrielle en France, comment pouvons-nous accepter de tels agissements ? Il paraît impensable que des entreprises inscrites au patrimoine vivant, qui s'impliquent pour développer le tissu économique de nos territoires et participent à l'excellence de notre rayonnement international soient mises de côté. Ce problème précis révèle une difficulté plus globale sur la commande publique et les appels d'offres qui ne mettent pas en place toutes les mesures possibles à l'attention des entreprises françaises, afin que celles-ci soient mieux prises en compte. Un appel d'offres devrait être très ouvert et, par exemple, ne citer que le type d'instrument de musique souhaité, sans indiquer une quelconque marque. Madame la ministre,

et les EPCI pour leurs achats. Des principes fondamentaux doivent être respectés : il en est ainsi de l'égalité de traitement qui prohibe toute pratique discriminatoire de nature à favoriser certains opérateurs, de la liberté d'accès qui permet à tout opérateur de se porter candidat, ou encore de la transparence des procédures. Si des illégalités ou des impropriétés ont été commises, il faudra remédier à ces manquements. Je souhaite cependant rappeler que, si les conservatoires sont classés par l'État, à la demande des collectivités, ils relèvent de l'initiative de celles-ci et de leurs responsabilités pleines et entières. La plupart des conservatoires sont ainsi gérés en régie directe et le principe de libre administration des collectivités territoriales ne permet pas à l'État de s'immiscer dans le fonctionnement de ces établissements, donc dans leurs politiques d'acquisition instrumentale. Pour ce qui concerne les évolutions à apporter à la commande publique- cela ne relève pas de mon

par le théâtre Bolchoï de Moscou, l'Opéra de Sydney, l'Orchestre philharmonique de Berlin et la Scala de Milan mais soient oubliés par l'Opéra de Paris

vous le savez, les sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué plus de vingt ans de service ont droit, à partir de 55 ans, au versement d'une rente annuelle appelée « Prestation de fidélisation et de reconnaissance », ou PFR. Le montant de cette prestation varie en fonction du nombre d'années de service ; il est fixé chaque année par arrêté ministériel. Pour tenter de contrer la baisse inquiétante du nombre de pompiers volontaires, une réforme de cette rente a été engagée par la loi du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires.

dans le Puy-de-Dôme, 89 dossiers sont encore en attente, ce qui retarde, parfois de plusieurs années, le versement de sommes pourtant largement méritées par des pompiers volontaires qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour la sécurité de tous. Les volontaires représentent 80 % des sapeurs-pompiers en France et constituent le socle de notre modèle d'intervention en matière d'incendie et de secours d'urgence aux personnes.

du statut des sapeurs-pompiers volontaires et par une protection sociale renforcée et adaptée. C'est dans cet esprit que la loi du 27 décembre 2016 précitée et le décret du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires ont créé la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, la NPFR, qui se substitue, depuis janvier 2016, à la prestation de fidélisation et de reconnaissance, la PFR, instituée par la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004. Il s'est agi d'une avancée sociale majeure, dont la mise en oeuvre, aujourd'hui achevée, donne entièrement satisfaction. Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1 janvier 2016 continuent de bénéficier l'ancien dispositif, qui était un régime de versement de prestations de fin de service par capitalisation. Cet ancien régime, qui prévoyait l'acquisition de points en fonction de seuils d'ancienneté d'activité des sapeurs-pompiers volontaires, pose aujourd'hui des difficultés à certains anciens sapeurs-pompiers volontaires, notamment lorsque des anomalies existent dans leur déroulé de carrière ou dans le versement de leurs cotisations. En effet, le régime étant clôturé depuis le 1 janvier 2016, à la suite de la création de la NPFR, aucun nouveau droit ne peut être créé sur les dossiers existants. Après une première phase de dialogue entre l'Association pour la PFR, chargée de ce régime, et CNP Assurances, gestionnaire du contrat, 282 dossiers en souffrance ont été régularisés en 2019. Ce dialogue s'est poursuivi,